son bébé, né avec le cordon ombilical autour du cou, est sain et sauf. Cette jeune mère avait une heure et quart de route à parcourir pour rejoindre la maternité de Périgueux, car celle de Sarlat, près de laquelle elle réside, ne pratique plus d’accouchements depuis le mois d’octobre 2024. L’histoire de cette femme n’est malheureusement pas un D’autres jeunes mamans ont récemment fait la une des journaux pour avoir accouché dans leur voiture, dans leur salon, voire dans un camion de pompiers. En cinquante ans, les trois quarts des maternités françaises ont disparu, à l’instar de celle de Sarlat, entraîne des accouchements extrahospitaliers et des risques accrus pour les femmes et les nourrissons. Il est prouvé que la mortalité néonatale est presque quatre fois plus élevée lorsque l’accouchement a lieu en dehors d’une maternité ou à plus de quarante cinq kilomètres de l’établissement le plus proche. Entre 1997 et 2019, le nombre de femmes en âge de procréer vivant à plus de quarante cinq minutes d’une maternité a plus que doublé. Alors que notre pays connaît une stagnation inquiétante de la mortalité infantile, la Cour des comptes préconise pourtant de poursuivre la fermeture des petites maternités. Ces fermetures renforcent le sentiment d’abandon des territoires ruraux, qui subissent déjà la désertification des services publics. Alors même que le Président de la République a appelé de ses vœux un « réarmement démographique » du pays, des territoires entiers se retrouvent dans des déserts obstétricaux et de nombreuses femmes vivent la fin de leur grossesse avec la peur de devoir accoucher dans leur voiture. En réalité, sous prétexte d’un impératif de sécurité, on les met en danger alors que nous manquons de praticiens, ces décisions de fermetures ne font que pousser les gynécologues à fuir. Madame la ministre, qu’envisage le Gouvernement pour revenir sur cette vision purement comptable et administrative de la question, qui nuit au maillage de l’offre de soins et à la sécurité des mères et des enfants à naître ?

L’accès à une prise en charge périnatale de qualité en tout point du territoire est un sujet d’attention particulière du Gouvernement, alors que les maternités, comme l’ensemble des activités des établissements de santé, connaissent aujourd’hui des tensions, liées principalement aux effectifs des soignants.

qui peuvent notamment fragiliser les petites maternités, ne constituent pas un obstacle à l’accès des femmes enceintes à une prise en charge sécurisée de leur grossesse, le plus près possible de leur domicile. Lorsqu’une maternité n’a pas d’autre choix que de fermer ses portes, faute de personnel disponible, l’agence régionale de santé (ARS) compétente se mobilise en lien avec les acteurs locaux pour mettre en place un ensemble de mesures

et de leurs nouveau nés. En outre, sur le site de l’ancienne maternité, des centres périnatals de proximité prennent alors le relais, pour offrir un panel large de soins en matière de périnatalité ; c’est absolument essentiel, alors que l’on constate, vous l’avez rappelé,

certains résidents au sens de l’Insee peuvent ne pas être des assurés sociaux français et inversement. En voici les raisons. Les bases qui permettent de décompter ces deux catégories de population n’intègrent pas des informations comparables ; surtout, elles ne visent pas les mêmes finalités. D’une part, le fichier de l’Insee recense les populations résidentes au terme d’une estimation statistique, après une collecte de données étalée sur cinq ans. D’autre part, le répertoire national inter régime des bénéficiaires de l’assurance maladie est une base de données qui permet la gestion des droits à l’assurance maladie, pour identifier les assurés sociaux et leur rattachement à l’assurance maladie. Ainsi, les assurés qui sont recensés n’ont pas forcément de droits ouverts à l’assurance maladie. Par exemple, les personnes décédées ou celles dont les droits sont fermés pour d’autres raisons, départ définitif à l’étranger, demeurent inscrites dans ce répertoire pour une durée maximale de deux ans. En revanche, leurs droits sont bien fermés dans les bases de gestion des caisses primaires d’assurance Pourquoi en est il ainsi ? La conservation de l’information du rattachement d’un assuré est nécessaire pour des raisons opérationnelles. Par exemple, des dépenses d’assurance maladie peuvent être traitées jusqu’à deux ans après le décès de la personne concernée ou à la fin de ses droits. Il est normal que les comptes de personnes décédées ne soient pas immédiatement supprimés, sans quoi les prestataires de santé seraient fortement pénalisés. L’assurance maladie a toutefois conduit un important travail de mise à jour des fins de droit dans le Rniam. Veuillez conclure,

aux soins. Madame la ministre, ma question devait initialement porter sur l’absence de publication de l’arrêté interministériel encadrant les nouvelles modalités de calcul du Nutri score. Elle est aujourd’hui caduque, car cet arrêté a enfin été publié. Cette mise à jour, fondée sur les dernières avancées scientifiques, permet de mieux prendre en compte la qualité nutritionnelle des aliments ultratransformés, trop gras, trop salés

donc : un blocage au bénéfice de qui ? Certainement pas des consommateurs, qui attendent une information plus fiable sur les aliments qu’ils consomment. Certainement pas non plus des entreprises qui jouent la transparence et qui essaient d’être plus vertueuses.

et mette tout en œuvre pour rendre le Nutri score obligatoire. Chaque recul face aux intérêts privés sape la crédibilité de nos institutions et freine des mesures pourtant essentielles pour la santé publique. Quelles garanties Quelles garanties donnez vous aujourd’hui pour que ces pressions n’entravent plus jamais les politiques de santé publique ? Quand la santé des Français passera t elle enfin avant les intérêts des géants de l’industrie ? La parole est à Mme la ministre.

a mené une évaluation complète des modalités de calcul du système, pour proposer des évolutions fondées sur des données scientifiques et des contributions des parties prenantes. Les évolutions prévues pour cet arrêté permettent notamment d’améliorer la différenciation entre les aliments selon leur teneur en sel et en sucre, et la riches en fibres et leurs substituts raffinés ou transformés. Elles améliorent en outre la classification des poissons gras et des huiles moins riches en acides gras saturés, ainsi que la différenciation entre les boissons selon leur teneur en sucre, tout en prenant en compte la présence d’édulcorants, afin de limiter leur usage en substitution du

et de l’emploi. Madame la ministre, les missions locales jouent un rôle essentiel dans nos territoires, crucial pour l’accompagnement social et professionnel des jeunes de 16 à 25 ans. Elles permettent le déploiement de politiques déployées par le tissu local, mais surtout la mise en œuvre de dispositifs de l’État, en premier lieu le contrat d’engagement jeune. Ce dispositif, dont le déploiement s’est accompagné de financements supplémentaires en direction des associations, a conduit ces dernières à recruter de nouveaux collaborateurs pour répondre à l’augmentation du nombre de bénéficiaires accueillis et accompagnés. À ce stade, les missions locales normandes n’ont pas de confirmation précise sur les financements de l’État pour l’année 2025, à l’exception d’une information transmise par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) de Normandie, qui leur a annoncé une éventuelle baisse de 5,9 % de leur dotation. Cette situation place les missions locales normandes dans une incertitude qui complique la planification de leurs actions et menace la pérennité de leurs missions. De plus, cette baisse intervient dans un contexte de hausse du taux de chômage des jeunes en Normandie. Au troisième trimestre de 2024, ce taux a atteint 7,2 %, ce qui représente une augmentation de 8,3 % du nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans sur un an. Dans ce contexte, il paraît crucial de renforcer les actions des missions locales, qui anticipent une augmentation du nombre de jeunes accueillis cette année.

le sénateur, je vous confirme que ces versements ont pu être réalisés à la fin du mois de mars, ce qui a permis de sécuriser la trésorerie des missions locales en début de gestion.

Malgré des indicateurs alarmants, ces établissements restent financièrement fragiles, surtout depuis la crise du covid 19. Dans ce contexte déjà tendu, un plan de 590 millions d’euros a été lancé, avec des investissements importants, comme la reconstruction de l’hôpital du Raincy Montfermeil. Toutefois,

Les conséquences sont déjà visibles : à Aulnay sous Bois, le service de diabétologie a fermé, alors qu’il répondait à un besoin crucial chez les plus modestes. Les syndicats hospitaliers, notamment la CGT 93, tirent la sonnette d’alarme depuis plusieurs mois. Ils dénoncent ce projet comme étant une régression sociale, tant pour le personnel que pour les usagers, et appellent à une réponse de l’État fondée sur l’égalité républicaine, non sur une logique purement comptable. Madame la ministre, quelles garanties pouvez vous apporter pour que la transformation du service hospitalier ne se traduise pas mécaniquement par des suppressions de services, par une perte d’attractivité pour les professionnels et, à la fin, par un recul de l’accès aux soins pour les habitants ?

en capital à hauteur de 339 millions d’euros et un autofinancement de 21 millions d’euros par cession. Des aides régionales en exploitation sont également mobilisées pour un montant de 47 millions d’euros, afin de sécuriser la trésorerie.

Face à cette tragédie, au lieu de se replier dans la douleur comme tant d’autres, il a fait le choix de l’action, en créant l’association Victimes du covid 19, dont l’objectif est d’honorer la mémoire de ceux qui ont succombé au virus et d’offrir à leurs proches un lieu de recueillement. Depuis lors, à Cormontreuil – sa commune –, mais aussi à Châlons en Champagne ou, plus récemment, à Taissy et à Reims, cet homme de 73 ans s’est engagé sans relâche pour convaincre les collectivités de mettre en place des lieux de mémoire : stèles, arbres, plaques commémoratives. Chaque installation a donné lieu à des hommages locaux, empreints d’émotion et de dignité. Aujourd’hui, je souhaite appeler votre attention sur son combat et sur la nécessité de prévoir un hommage national à la mémoire des victimes de la pandémie de covid 19, une crise qui a profondément marqué notre pays. Rappelons nous : le 17 mars 2020, la France est entrée dans un premier confinement strict, bouleversant le quotidien de tous nos concitoyens. Cette date, devenue le symbole d’un bouleversement sanitaire, social et humain sans précédent, marque cette année son cinquième anniversaire. Durant cette période sombre, des milliers de familles ont été endeuillées, souvent dans des conditions particulièrement cruelles : sans adieux, sans cérémonie, sans possibilité d’accompagner leurs proches dans leurs derniers instants. Au delà de la souffrance causée par la maladie, l’isolement dans la mort et la privation de rituels essentiels au deuil ont laissé des cicatrices profondes. Aujourd’hui encore, beaucoup ressentent le besoin d’un moment de reconnaissance collective, d’un temps de mémoire pour apaiser les douleurs et tourner une page douloureuse de notre histoire commune. Certes, d’autres urgences occupent désormais l’agenda politique, mais il paraît indispensable qu’un hommage national puisse être institué, afin que la Nation dans son ensemble puisse se recueillir. Un tel moment, empreint de solennité et de respect, permettrait non seulement d’honorer les disparus, mais aussi d’apporter un soutien symbolique aux familles qui restent. Il s’agirait non de rouvrir les débats ou les polémiques, mais d’affirmer l’importance du devoir de mémoire, du lien entre les générations et de notre capacité à nous rassembler dans les épreuves.

Monsieur le sénateur Cédric Chevalier, votre question nous rappelle que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle des chocs externes : crises

un geste fort de la République. Un hommage solennel, inscrit durablement dans notre calendrier républicain, serait un acte de reconnaissance, d’unité et de résilience nationales. Il pourrait rassembler autour de notre histoire récente nos douleurs partagées et, surtout,

Ces délais de traitement excessifs résultent de moyens notoirement insuffisants. Pour fonctionner correctement, la structure devrait compter quinze médecins ; or ils ne sont que Des opérations « coup de poing » ont été menées pour absorber les dossiers en attente, au détriment des rendez vous et des visites à domicile. Forcément, la satisfaction des usagers a chuté, passant de 70 % en 2022 à 44 % en 2023. En outre, les conditions de travail du personnel se dégradent.

Madame la sénatrice Aeschlimann, depuis leur création en 2006, les MDPH ont vu leur activité tripler.

rapport à 2022. Le nombre de postes budgétaires a connu, parallèlement, une augmentation progressive, mais les recrutements sur les postes vacants restent difficiles. L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, qui représente 59 % des postes budgétaires, est particulièrement touchée par ces difficultés de recrutement.

à leur mission. Dans un jugement du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a considéré que le courrier envoyé par un assistant familial dans lequel celui ci ne renonce qu’à son agrément ne peut être considéré comme une lettre de démission.

d’une rupture du contrat de travail sur l’initiative de l’employeur, qui ouvre droit aux indemnités. Face aux demandes de plus en plus fréquentes de ce type, les départements ont deux options : soit ils refusent la demande de retrait de l’agrément, au risque de mettre en péril

présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; passer un examen médical ayant pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d’accueillir habituellement des mineurs ; disposer d’un logement. Si ces conditions ne sont plus remplies, le président du conseil départemental peut procéder au retrait de l’agrément après avis de la commission consultative. Cette décision doit être motivée et collégiale, et elle est susceptible de recours. L’assistant familial qui fait l’objet d’un retrait d’agrément ne peut plus exercer sa profession et ses employeurs doivent alors le licencier. alors le licencier. Le souhait d’un assistant familial de se voir retirer son agrément ne constitue pas un motif légitime de retrait d’agrément. L’assistant familial ne peut être à l’initiative d’un retrait d’agrément, et il ne peut être mis fin au contrat que par rupture conventionnelle ou par démission.

de notre système de protection de l’enfance. Je pense d’abord au procès du drame d’Amandine, jeune fille de 13 ans morte de faim et à la suite des mauvais traitements infligés par sa mère. Comment un tel drame a t il pu se produire malgré les signalements répétés aux services sociaux ? Pourquoi l’État n’a t il pas pu ou su protéger cette enfant ?

En octobre 2024, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a confirmé ce diagnostic alarmant. Le 28 janvier dernier, la Défenseure des droits a également dénoncé la dégradation préoccupante de la protection de l’enfance, soulignant que cette situation portait atteinte à l’intérêt supérieur et aux droits fondamentaux des enfants. Près de 400 000 mineurs ou jeunes majeurs sont pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE), mais celle ci peine à leur apporter la protection et l’aide nécessaires. Quelque 30 000 postes sont vacants dans les établissements du secteur médico social, et 70 % des juges interrogés déclarent avoir déjà renoncé à placer des enfants faute de solution adéquate. En outre, l’accès aux soins n’est pas pleinement garanti. Les départements, étranglés financièrement par les baisses de dotations et les transferts de charges non compensés, peinent à assumer leurs responsabilités en la matière. La responsabilité de l’État, qui ne dispose même plus d’un ministère de plein exercice dédié à cette cause, est flagrante. L’obsession sécuritaire à l’encontre des mineurs a pris le pas sur la responsabilité de protéger les plus faibles, en particulier les enfants.

Dans le domaine de la santé, un bilan psychologique et somatique sera systématiquement réalisé dès la prise en charge des enfants, conformément au souhait de Mme Vautrin. Le placement à dimension familiale doit être privilégié pour offrir aux enfants un environnement stable et chaleureux.

parcours emploi compétences » (PEC) au sein des collectivités territoriales. Depuis le 1 janvier 2018, les contrats aidés dans les collectivités et associations ont été transformés en PEC, afin de faciliter l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi. Pour des milliers de

concernent des milliers d’agents d’accueil, de restauration scolaire, de service technique, qui agissent au plus près des habitants. Ils constituent donc un outil majeur pour les collectivités territoriales, notamment rurales, dont les marges de manœuvre sont financièrement restreintes, alors que les besoins de service public n’ont jamais été aussi importants. Malgré cela, on constate depuis plusieurs années une réduction significative du nombre de contrats PEC à l’échelle nationale.

Madame la ministre, le maintien du nombre de PEC étant indispensable pour assurer la continuité des services publics, quelles mesures le Gouvernement envisage t il de prendre pour soutenir les collectivités territoriales face à l’annonce de leur réduction brutale et sévère ? La parole est à Mme la ministre.

Si les détenus bénéficient systématiquement d’escortes sécurisées lors de consultations hospitalières conventionnelles, il n’en va pas de même lorsqu’ils présentent des troubles psychiatriques nécessitant une hospitalisation. un arrêté de soins sans consentement sur décision d’un représentant de l’État (SDRE), le préfet détermine la nature de l’escorte et, force est de le constater, les soignants sont très fréquemment contraints contraints d’assurer le transport de ces patients, s’exposant ainsi à des risques majeurs pour leur sécurité. En outre, en cas d’hospitalisation, un transfert de responsabilité s’opère entre le directeur de l’établissement pénitentiaire et celui du centre hospitalier. Le détenu devenu patient patient dispose de droits régis par le code de la santé publique et non plus par le code pénitentiaire. Néanmoins, aucune information relative à la nature de la détention ou à la dangerosité des individus n’est communiquée aux personnels de santé.

Monsieur le sénateur Franck Menonville, vous m’interrogez sur la sécurité des soignants au contact de détenus qui nécessitent un suivi psychiatrique. Dans le cadre de la dernière feuille de route Santé des personnes placées sous main de justice, une action est consacrée à « l’amélioration du parcours de soins en santé mentale sur […] trois niveaux ». Vous le savez, bien que la

à prendre en charge des patients détenus, en apportant des réponses concrètes à chacune des difficultés rencontrées. Il rappelle notamment les règles applicables en matière d’escorte, ainsi que les modalités d’application des droits fondamentaux des patients. Parallèlement, le ministre de la santé copilote avec le ministre de la justice le déploiement de la seconde tranche des UHSA, avec la construction de trois nouvelles unités. Celles ci permettront la création de 160 lits supplémentaires, s’ajoutant aux 440 lits déjà existants. Enfin, il faut souligner les travaux parlementaires

et numérique, chargée des comptes publics. la ministre, en 2018 était signée la nouvelle convention fiscale entre la France et le Luxembourg. Son objectif était simple : éviter la double imposition, mais aussi lutter contre la fraude fiscale. Elle a été amendée à deux reprises, et son entrée en vigueur a été repoussée d’autant depuis sa signature. Le ministre de l’époque, M. Bruno Le Maire, s’était engagé à effectuer une étude d’impact afin de mesurer ses effets sur le taux d’imposition des ménages concernés. Dernièrement, le Gouvernement a annoncé appliquer les dispositions de la convention fiscale sur les revenus faisant naître de vives inquiétudes dans nos territoires. En effet, les conséquences de cette réforme pour les contribuables frontaliers, particulièrement pour les retraités et ceux qui disposent de revenus mixtes, seraient loin d’être neutres.

Néanmoins, le passage d’une méthode à l’autre pourra avoir une incidence sur le taux d’imposition appliqué en France sur les autres revenus perçus en France. La méthode précédemment utilisée limitait la progressivité de l’impôt appliqué aux revenus imposables en France. Sur ce point,

que ceux des foyers qui, à montants équivalents, ne disposent que de revenus de source française. Il s’agit donc d’une réforme d’équité. L’application pleine et entière de la convention permettra donc de rétablir l’égalité de traitement des frontaliers et des autres résidents.

2024. Le projet d’Accolans a été déposé antérieurement à la publication du décret du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles,

en février 2025 pour clarifier la trame devant être suivie par les services instructeurs. Nous restons donc pleinement à l’écoute des différents acteurs afin de lever les barrières au développement d’un agrivoltaïsme raisonné, qui doit reposer sur de la confiance de la stabilité. Nous laissons évidemment de la place à l’innovation technologique pour accompagner les projets. Les services instructeurs disposent aujourd’hui de tous les éléments pour prendre

Madame la ministre, la souveraineté et les ambitions énergétiques de la France sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens et des élus dans les territoires.

Depuis une décennie, la France résiste à l’ouverture à la concurrence. Le soutien politique transpartisan en la matière signe la volonté de maîtriser notre souveraineté énergétique.

L’enjeu est d’autant plus important que les barrages contribuent à atténuer les pénuries d’eau et à prévenir les inondations en régulant les flux, grâce à une gestion plus adaptée et plus concertée qu’auparavant.

Aujourd’hui, nous avons le sentiment d’être dans une impasse, au point mort, bloqués dans un précontentieux avec la Commission européenne. Chaque partie s’accorde sur la nécessité de moderniser les installations hydroélectriques, de conforter l’industrie de l’hydroélectricité et de maintenir les compétences dans ce domaine. C’est le cas de la Commission européenne, qui a publié à la fin du mois de février dernier un rapport sur la compétitivité des technologies énergétiques propres. C’est le cas également du Gouvernement puisque la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie, soumise à consultation publique jusqu’à la mi avril 2025, prévoit d’augmenter les capacités de la grande hydroélectricité. Reconnaissez, madame la ministre, que, sans visibilité et sans stabilité pour les exploitants, cette ambition sera vaine

de 2,8 gigawatts à l’horizon 2035. Les enjeux de l’usage de l’eau seront également déterminants pour l’alimentation en eau potable, l’irrigation et le soutien d’étiage. Or, vous l’avez dit, nous nous trouvons dans une situation de contentieux avec la Commission européenne

Il concerne les contribuables français ayant des revenus de source mixte, française et luxembourgeoise. Je tiens à rappeler les engagements pris par M. Bruno Le Maire : il avait assuré que ce nouveau mode n’aurait aucune conséquence financière pour les contribuables concernés et que cette réforme serait précédée d’une étude d’impact

à une étude d’impact. Des cas concrets de hausses d’imposition m’ont été rapportés par les contribuables concernés. Après discussion avec le cabinet de M. le ministre de l’économie, il semble que cette évolution

Cette double imposition est une violation manifeste de l’accord qui lie nos deux pays. Malgré des mois de démarches et de promesses de traitement du dossier par les autorités françaises, rien n’a changé depuis désormais Pis, la situation s’aggrave. Ces salariés reçoivent relance sur relance du fisc espagnol, la dernière datant du 10 mars dernier. Des intérêts de retard leur sont même désormais réclamés ! L’administration française est pourtant informée depuis longtemps de cette situation. Une procédure amiable a été ouverte, un moratoire annoncé et une réunion avec les autorités fiscales espagnoles prévue

je vous remercie

ayant une résidence fiscale en France et un domicile situé à moins de vingt kilomètres de la frontière. L’administration fiscale leur réclame le paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques en Espagne et considère qu’ils ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal des travailleurs transfrontaliers, situation qui conférerait le droit d’imposition à la France.

Néanmoins, mes services, la direction de l’hôpital et les salariés sont dans leur bon droit de considérer que cet article ne s’applique pas à une personne morale partagée par les deux États, telle que l’hôpital de Cerdagne, qui est, comme vous l’avez dit, un groupement européen de coopération territoriale. Saisi de la situation par les intéressés et en lien avec la direction de l’hôpital, le service chargé de la résolution des différends internationaux de la DGFiP, qui se trouve sous mon autorité, a pris attache avec son homologue espagnol afin de trouver au plus vite une solution une solution à cette situation que je qualifierai d’inacceptable. Il est important que nous prenions en compte les discussions qui ont déjà eu lieu entre les administrations fiscales française

Néanmoins, à ce jour, il subsiste toujours une divergence profonde dans l’analyse du régime applicable. La situation de blocage ayant été constatée sur le plan administratif, il a été décidé que cette question serait portée au plus haut niveau. Notre ambassadrice à Madrid écrira prochainement à la ministre des finances espagnole

pris en application de l’article L. 34 9 1 du code des postes et des communications électroniques impose aux opérateurs de téléphonie mobile de transmettre un dossier d’information mairie (DIM) à la collectivité concernée. L’objectif est d’informer la municipalité du projet d’installation faciliter ainsi l’instauration d’un dialogue entre les élus et les habitants de la commune. Toutefois, l’autorisation d’urbanisme n’étant pas conditionnée au dépôt du dossier d’information mairie, une déclaration préalable de travaux peut être acceptée quand bien même la mairie n’aurait pas encore eu connaissance du projet d’implantation. Aussi, découvrant ce projet au dernier moment, les élus ne sont plus en mesure d’informer et de consulter leurs administrés dans de bonnes conditions, créant ainsi incompréhension et frustration de part et d’autre. Pourtant, le développement du réseau mobile reste un enjeu majeur dans les zones rurales. Madame la ministre, dans un contexte où les maires ont besoin de retrouver de la capacité d’action,

Il est extrêmement important aussi que nous vérifiions la conformité de l’antenne aux valeurs limites d’exposition du public aux ondes et l’absence de brouillage préjudiciable aux autres utilisateurs, ce que vérifie l’ANFR. le sénateur, il n’y a ni incohérence de la réglementation ni dépossession des maires de leur pouvoir de police. Le processus est garant du respect des valeurs d’exposition du public aux ondes. Nos concitoyens peuvent être rassurés sur ce point. Toutefois, certaines difficultés sont remontées par les élus locaux. C’est d’ailleurs pour cela que le Gouvernement avait proposé dans la version initiale du projet de loi de simplification de la vie économique un droit pour les maires de ne pas revenir sur une décision favorable ou de non opposition à l’implantation d’une antenne relais.

et que les opérateurs sollicitent fréquemment un délai plus court. Je suis pour ma part très attachée à ce que tant les élus locaux que la population soient informés dans de bonnes conditions, gage d’acceptabilité

par une fraction de l’accise sur l’électricité, cette mesure remet en question un mécanisme de financement historique des syndicats d’énergie, menaçant leur capacité à financer les investissements dans les zones rurales. Au lieu de simplifier le système, cette réorganisation pourrait entraîner une réduction importante des investissements en faveur de la transition énergétique et de la prévention des aléas climatiques, particulièrement dans les communes rurales, déjà confrontées à une diminution de leurs financements. les répercussions ne se limiteraient pas à une dégradation du service public. Elles représenteraient également une véritable menace pour l’économie rurale, qui repose sur des infrastructures énergétiques fiables et résilientes.

Derrière l’objectif affiché de simplification, c’est en réalité l’existence même du CAS Facé qui est menacée, car la réforme déconnecte le financement des réseaux des besoins réels et accentue les disparités entre zones rurales et zones

En ce qui concerne les modalités d’attribution des aides, elles demeurent inchangées dans cette loi de finances : la répartition des dotations entre départements n’est ainsi pas modifiée et les dossiers de demande de subvention continueront d’être instruits comme précédemment. Parce que nous savons que l’électricité joue un rôle déterminant dans le quotidien des Français et de nos entreprises, le Facé continuera à être une politique structurante dans les territoires ruraux afin de leur garantir une électricité de qualité. C’est un gage de cohésion entre les territoires urbains et ruraux. Ce compte fait partie intégrante du service public de l’électricité

J’ai été alerté sur des dérives graves : soupçons de corruption, délivrance illégale de grades, opacité financière, verrouillage des élections internes. De plus, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a établi un constat sans ambiguïté concernant l’élection à la présidence de la Fédération, qui avait cristallisé l’ensemble des alertes et des critiques. Pour sortir de cette crise, le CNOSF a recommandé l’organisation d’un nouveau scrutin, proposition que la présidence de cette fédération a refusée.

Madame la ministre, 250 000 licenciés attendent aujourd’hui que l’État se tienne à leurs côtés. L’héritage des jeux Olympiques ne saurait être ni à géométrie variable ni à la carte. Cet héritage, c’est aussi le respect des règles, à tous les niveaux

qui est de l’assemblée générale élective du 12 décembre 2024, vous l’avez dit, la conférence des conciliateurs du CNOSF, dans son avis, a reconnu l’inégalité de traitement entre les candidats et a préconisé l’organisation de nouvelles élections à la présidence. M. Bruno Verfaillie, le président élu, a refusé cette proposition de conciliation. Les opposants ont désormais la possibilité de contester cette

La Fédération française de karaté et disciplines associées est citée dans cette procédure pour avoir perçu des fonds liés à la liquidation de la zone interdépartementale Dauphiné Savoie. Les conclusions du parquet n’ont pas encore été communiquées, l’enquête étant toujours en cours.

lui sera alors retiré. La FFKDA a en outre été auditionnée le 5 juillet 2024 dans le cadre de la mission d’inspection générale sur les sports de combat diligentée sur l’initiative

Rassemblant aujourd’hui près de 200 cercles celtiques et 15 000 adhérents, elle peut se prévaloir d’un rayonnement dépassant largement les frontières régionales. Reconnue par l’éducation nationale comme association complémentaire de l’enseignement public et par les collectivités bretonnes comme structure d’enseignement artistique et culturel,

La condition stricte exigeant que les projets soient portés par des chorégraphes professionnels ayant diffusé des pièces dans le « réseau » de danse prive la confédération de l’accès au financement de la CDC, alors

Ce refus est le symptôme d’un problème plus large : l’insuffisance du soutien de l’État et de ses opérateurs à la valorisation de la « matière culturelle bretonne » et à ses acteurs, qui jouent pourtant un rôle déterminant dans le bien vivre ensemble et dans la transmission et la vitalité de notre patrimoine immatériel, et ce sur l’ensemble du territoire régional, notamment rural. Cette carence concerne aussi la transmission de la musique : elle affecte notamment les, ces ensembles musicaux emblématiques de la culture bretonne, rassemblés au sein de la confédération Sonerion,

Alors que la direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Bretagne reconnaît l’utilité publique de la confédération Kenleur et l’accompagne le dispositif d’aide au service des publics, comment justifier que la Caisse des dépôts et consignations, qui est sous tutelle de l’État, n’en fasse pas de même ?

Mme la ministre. Monsieur le sénateur Uzenat, les arts et traditions populaires sont source de lien social ; ils témoignent de la grande diversité culturelle de nos territoires. Pourtant, comme vous l’avez rappelé, ces pratiques ont souvent été l’angle mort de nos politiques culturelles.

aux musiques et danses traditionnelles, ainsi qu’aux pratiques inscrites au patrimoine culturel immatériel, comme le en Bretagne. La Drac de Bretagne y est très attentive. Elle a notamment noué des relations étroites avec la confédération Kenleur, qu’elle soutient dans le développement de ses différentes actions un festival d’été itinérant permis par le dispositif « Été culturel », ou encore les manifestations financées en ruralité dans le cadre des « Villages en fête ». Au total, en 2024, la confédération Kenleur a ainsi bénéficié de 40 500 euros d’aides aux projets de la part de la Drac.

ar Sonerion ; des équipes artistiques, comme la compagnie de danse C’hoari ; des lieux de diffusion, comme La Grande Boutique ; des structures de valorisation de la culture et de l’identité bretonnes, comme l’association Bretagne Culture Diversité. Soyez convaincu, monsieur le sénateur, que le ministère de la culture suit de près la situation de la confédération Kenleur. La parole est à Mme Mireille Jouve,

Il bataillait sans relâche sur le dossier des aménités rurales, en sa qualité de président du grand site Concors Sainte Victoire. Les aménités, c’était son sujet ; c’est notre sujet. Comme nombre de maires ruraux, il était inquiet de la révision des critères d’éligibilité à la dotation

Les maires ne sauraient se satisfaire de la note d’information qui leur a été communiquée le 11 juillet dernier : la réforme, y est il écrit, « vise à reconnaître et valoriser davantage les services environnementaux rendus par les communes rurales à l’ensemble de la Nation en termes de maintien des réservoirs de biodiversité ».

et la ruralité à habitat très dispersé. Ce critère a conduit à ne plus prendre en compte 146 communes qui percevaient la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales mise en place en 2019. Il a également conduit à prendre en compte 2 680 communes qui n’y étaient pas éligibles en 2023, 8 921 communes rurales étant éligibles à la dotation en 2024. Sont intégrées au dispositif l’ensemble des communes dont une part importante du territoire est consacrée à la protection de la biodiversité, en cohérence avec la stratégie nationale des aires protégées, et non plus seulement les communes situées en parc national, en parc naturel marin ou en site Natura 2000. de la dotation passe ainsi de 41,6 millions d’euros à 100 millions d’euros entre 2023 et 2024. Cette réforme concourt ainsi au double objectif de reconnaître la contribution des communes rurales

à couvrir le territoire national de 30 % d’aires protégées bien gérées et de 10 % d’espaces sous protection forte. Enfin, la dotation n’est pas le seul outil de valorisation de l’engagement des collectivités

produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB). Or de graves manquements m’ont été signalés, qui s’accumulent depuis la création de l’entreprise en 2012, tant en matière de respect du droit du travail que de respect des normes environnementales. En septembre 2024, plusieurs salariés ont exercé leur droit de retrait après des contrôles positifs à l’amiante. Depuis des années, l’entreprise n’offrirait ni protection ni formation adéquate à ses employés, exposant de surcroît les riverains à des poussières potentiellement toxiques. Les cartons jaunes se sont succédé, mais, malgré des constats d’irrégularité dressés de manière répétée par l’inspection des installations classées, l’entreprise poursuit ses activités sans entrave notable.

partie du plâtre sortant de l’entreprise contienne de l’amiante et soit réintroduit sur le marché sans contrôle adéquat. En outre, la liberté syndicale et le droit des lanceurs d’alerte sont

protéger les travailleurs exposés à l’amiante, ainsi que les riverains et l’environnement, et garantir un recyclage réellement sûr et responsable

Ainsi, depuis 2022, trois mises en demeure ont été adressées à l’exploitant de ce site et deux amendes administratives ont été prononcées par le préfet à la suite de constats de non conformité persistants. Dans le cadre d’un contrôle engagé depuis plusieurs mois, l’inspection du travail a par ailleurs rappelé à l’employeur les principes généraux de prévention et l’obligation générale de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs. Elle a demandé que des mesures adaptées soient prises afin d’assurer la protection des salariés, notamment en ce qui concerne leur exposition aux émissions de poussières et à l’amiante. Ce contrôle se poursuit et l’entreprise fait l’objet d’un suivi spécifique de la part de l’inspection du travail. viens à la filière à responsabilité élargie des producteurs des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. L’entreprise Ritleng Revalorisations est en effet l’un des prestataires de l’éco organisme agréé Valobat.

des chantiers et des centres de massification des déchets avec lesquels il est en contrat. Par ailleurs, en application du code de l’environnement, l’éco organisme Valobat a conçu un programme d’audit auprès de ses prestataires gérant des déchets.

que fait peser cette réforme sur l’emploi des marins français, sur le maintien de notre pavillon et sur notre place dans la transition écologique maritime. Cette hausse soudaine des coûts d’exploitation de 25 provoque un surcoût non budgété de 2,2 millions d’euros pour les armateurs havrais. Elle met en péril leur modèle économique. L’entreprise Towt est particulièrement affectée alors qu’elle développe un transport français à la voile relevant pleinement Elle prévoyait, d’ici à 2027, la mise en service de six nouveaux voiliers cargos, en plus des deux déjà existants, Artemis et Anemos. De même, l’entreprise Sogestran, spécialiste du transport fluvial, qui a baptisé son premier navire à hydrogène, est fortement touchée,

Mme la ministre. Madame la sénatrice Canayer, le secteur du transport et des services maritimes fait face à une intense concurrence internationale. La compétitivité des pavillons repose en grande partie sur les coûts salariaux, principal facteur discriminant par rapport aux autres coûts d’exploitation.

L’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 modifie la donne : depuis le 1 mars 2025, le bénéfice de la totalité des exonérations est réservé aux seuls armateurs opérant des navires de transport de passagers, des navires câbliers et des navires de service consacrés aux énergies marines renouvelables. En revanche, les autres segments de flotte perdent l’exonération des parts « chômage » et « famille », tout en conservant l’exonération des cotisations pour les gens de mer affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins. Il est à noter que cette dernière part, dite Enim, reste prépondérante au sein de l’ensemble des exonérations. Comme vous le savez, la situation financière du pays impose des choix budgétaires responsables. Comme d’autres, la mesure sur laquelle vous m’interrogez permet de réaliser des économies, contribuant ainsi à l’effort collectif de redressement des finances publiques. Nous mesurons toutefois combien les effets de cette réforme sont significatifs : plusieurs armateurs ont publiquement fait part de leur intention de changer de pavillon, notamment les entreprises de la filière vélique, ce qui témoigne des tensions suscitées par cette Conscients de ces signaux, nous avons d’ores et déjà prévu une évaluation approfondie du dispositif visant à en apprécier pleinement les effets économiques et budgétaires : il va nous falloir comparer les gains réalisés aux effets produits sur la compétitivité du pavillon français. Le cas échéant, et à la lumière de cette évaluation, le Gouvernement n’exclut pas de rouvrir le débat lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. La parole

suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ; les plombs de chasse seraient interdits dans un délai de trois ans ; la vente au détail des cartouches à plomb serait prohibée dans un délai de cinq ans.

de restriction de mise sur le marché pour les balles de plomb. L’usage des balles resterait autorisé dans les centres de tir, intérieurs comme extérieurs – ceux ci seraient toutefois soumis à autorisation préalable.

Si des subventions sont prévues le fonds Barnier, leur montant est insuffisant. Le plafond de 80 % des dépenses ne s’applique qu’aux dossiers validés avant 2027, contre un Ce calendrier est irréaliste compte tenu de la longueur des procédures administratives, de l’ampleur des travaux, de la nature des contraintes techniques et environnementales et de la disponibilité des entreprises. Pour le Sisarc, les quatre vingt dix kilomètres transférés nécessitent près de 110 millions d’euros hors taxe de travaux.

je vous remercie pour donner aux « Gemapiens » les moyens d’exercer leur compétence. La loi Maptam de 2014 avait prévu une période de transition de dix ans dans le cas des digues domaniales, qui représentent moins de 10 % des digues dans la France entière et dont l’État a poursuivi temporairement la gestion pour le compte des Gemapiens. période a pris fin le 28 janvier 2024. La très grande majorité de ces ouvrages a été reprise en gestion par les Gemapiens, par voie de convention. En Savoie, le syndicat mixte de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie s’est vu confier un linéaire d’ouvrages d’environ Des travaux de réhabilitation sont en cours, financés en totalité par le fonds Barnier, à hauteur de 6 millions d’euros. D’autres travaux prioritaires ont été programmés par le Sisarc, pour 46 millions d’euros ; le syndicat mixte les financera sans reste à charge

afin que le reste à charge, une fois optimisées les recettes procurées par la taxe Gemapi, soit aussi réduit que possible. Par ailleurs, compte tenu du rôle joué par ces ouvrages pour la protection d’infrastructures routières et ferroviaires stratégiques, d’autres contributeurs pourraient être appelés à soutenir leur financement à long terme. Enfin, l’obligation d’inscrire les ouvrages dans l’actif comptable de la collectivité est une mesure technique sans effets sur ses finances. La parole

De même, l’exploitation de la forêt paysanne favorise une filière locale de bois énergie bon marché et durable. Ce secteur économique dynamique regroupe notamment les fabricants, distributeurs et installateurs d’équipements de chauffage au bois.

Ces nouvelles normes pourraient avoir des effets considérables sur la filière, en contraignant les professionnels à revoir leurs gammes de produits et en obligeant les consommateurs à investir dans de nouveaux équipements. initialement être présentée le 12 février 2025, cette réforme a été reportée en raison des incertitudes sur sa faisabilité technique et économique. Ce report prolonge l’incertitude et les nombreuses interrogations des acteurs du secteur, l’attente de précisions sur les seuils retenus et sur les délais de mise en conformité. Les professionnels s’interrogent sur les adaptations techniques nécessaires pour répondre aux futures exigences. Quant aux ménages, ils redoutent les coûts élevés de remplacement ou de mise aux normes de leurs équipements. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’aucune solution de substitution réellement viable n’a été présentée. Afin d’éviter de fragiliser des milliers de foyers et de compromettre l’avenir de la filière du bois énergie, il importe qu’il n’y ait pas d’interdiction sans solution. pas d’interdiction sans solution. Dans ce contexte, madame la ministre, pouvez vous apporter des précisions sur le contenu de la future réforme et sur les dispositifs d’accompagnement qu’il conviendra de mettre en place pour soutenir les professionnels de la filière et les ménages concernés par ces évolutions réglementaires ? La parole

Le Gouvernement suit activement les travaux européens sur la réglementation relative à la mise sur le marché des équipements de chauffage au bois, qui vise à améliorer leur efficacité énergétique et à réduire leurs émissions de polluants atmosphériques, sans interdire leur installation ni imposer le remplacement des équipements existants. Cette réglementation simplifie l’accès au marché européen pour les fabricants, en uniformisant les normes pour toute l’Europe, tout en veillant aux bénéfices rendus aux utilisateurs. Les règlements, en vigueur depuis 2020, pour les chaudières fonctionnant à la biomasse, et depuis 2022, pour les poêles à bois, font l’objet d’une mise à jour. Celle ci a notamment pour objectif d’améliorer la réparabilité et la performance des nouveaux appareils, appareils, l’efficacité de leur consommation de combustibles et la réduction des émissions de polluants atmosphériques, sans interdire la conservation des équipements déjà installés. La Commission européenne a publié en janvier 2025 des documents de travail préliminaires afin de recueillir l’avis technique des experts et des parties prenantes. Une analyse de 14 000 produits vendus en Europe a déjà été réalisée

Le Gouvernement veillera à mettre en œuvre une approche équilibrée, conciliant exigences environnementales et réalités économiques, et accompagnera les professionnels et les ménages dans cette transition. La parole est à M.

à ce jour, aucune solution de remplacement n’est prévue pour les communes bénéficiaires. Pour rappel, ce fonds est subordonné à l’organisation au bénéfice des élèves scolarisés sur le territoire d’activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial et à une organisation du temps scolaire sur neuf demi journées ou huit demi journées comprenant cinq matinées. Ces aides sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles dans la commune et comprennent un montant forfaitaire ainsi qu’une majoration qu’une majoration forfaitaire en faveur des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine cible ou à la dotation de solidarité rurale cible. En Haute Vienne, quatre communes, Nieul, Peyrilhac, Saint Gence ont maintenu, dans le cadre du projet éducatif de territoire 2024 2027, l’organisation sur cinq matinées. le syndicat intercommunal enfance, petite enfance et adolescence, elles proposent une offre d’activités périscolaires de grande qualité à l’ensemble des enfants scolarisés. De surcroît, dans un souci de réduction des inégalités, les communes et le syndicat intercommunal ont fait le choix de les rendre gratuites pour tous. Madame la ministre, il est indispensable de préserver de tels services à la population et de soutenir les communes rurales qui les mettent en œuvre. Le Gouvernement va t il revenir sur la suppression du fonds de soutien aux TAP

vous l’avez rappelé, le fonds de soutien au développement des activités périscolaires avait pour objectif de contribuer à mettre en place des activités périscolaires lors du passage à une organisation scolaire sur quatre jours et demi. Ce fonds avait une durée limitée : la loi de 2013, qui l’a créé,

Il apparaît que le fonds n’incite pas les communes à maintenir la réforme des rythmes scolaires pour les élèves de leur territoire, raison pour laquelle son extinction a été programmée pour la rentrée 2023. Toutefois, répondant à l’inquiétude des élus, le Gouvernement a choisi de reporter son extinction pour permettre aux collectivités d’avoir le temps de s’adapter. Cette décision ne remettait cependant pas en question le principe de la suppression du FSDAP pour la rentrée 2025, qui a été acté dans la loi de finances pour 2024. Un nouveau report ne peut pas être envisagé, par la voie réglementaire. Enfin, dans un contexte budgétaire contraint, la ministre Élisabeth Borne a fait le choix de recentrer ces crédits sur d’autres dispositifs et d’autres priorités sociales. Je pense notamment aux crédits ouverts dans le cadre de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.

ministre déléguée. Monsieur le sénateur Pascal Savoldelli, plusieurs collectivités ont en effet pris la décision de mettre en place des autorisations spéciales d’absence (ASA) pour congé menstruel. Ces autorisations permettent ainsi, et c’est heureux, aux femmes souffrant de règles douloureuses, d’endométriose, d’adénomyose ou de dysménorrhées invalidantes de s’absenter de leur service, sans effet sur leurs droits à congés annuels. Toutefois, cette initiative soulève des questions juridiques importantes. En l’état actuel du droit, la création d’une nouvelle catégorie d’ASA pour raison de santé ne relève pas des compétences des collectivités locales. En effet, l’article L. 622 1 du code général de la fonction publique prévoit des autorisations spéciales d’absence pour des motifs spécifiques, tels que la parentalité ou certains événements familiaux, mais pas pour raison de santé. Ainsi, la mise en place d’un tel dispositif par les collectivités repose sur une base légale très contestable. C’est pourquoi le tribunal administratif de Toulouse a suspendu, le 20 novembre 2024, les délibérations de deux collectivités ayant instauré un congé menstruel, estimant que celles ci étaient incompatibles avec le droit, en l’absence, à ce jour, avec le droit, en l’absence, à ce jour, de dispositions législatives ou réglementaires permettant de le faire. Consciente de l’intérêt porté à cette question et de la demande croissante des collectivités et des administrations, la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) travaille actuellement à l’identification de solutions juridiques permettant de mieux prendre en compte ces situations, afin de leur apporter une réponse adaptée. La parole

collectivités locales et de leurs équipes se multiplient, ce qui soulève de nombreuses inquiétudes quant à la sécurité juridique des agents concernés. En effet, le champ des responsabilités des directions générales, bien que partiellement encadré par la loi, n’est pas encore suffisamment clair. La principale incertitude porte sur la notion de faute grave, qui n’est pas précisément définie dans l’ordonnance de novembre 2022. Lors d’une réunion sur la mise en œuvre de cette réforme, le président de la chambre du contentieux de la Cour des comptes, Serge Barichard, a précisé que cette notion serait progressivement clarifiée par la jurisprudence, tout en insistant sur le fait que seuls les manquements les plus graves donneraient lieu à des poursuites. Autrement dit, le champ des responsabilités sera affiné au fur et à mesure par les juges. Cette incertitude crée un climat d’insécurité pour les gestionnaires publics, qui doivent exercer leurs missions sans cadre précis leur permettant d’anticiper d’éventuelles mises en cause. Par ailleurs, dans sa décision du 29 janvier 2025, le Conseil d’État a rappelé que la protection fonctionnelle s’appliquait aux agents publics poursuivis pénalement. Toutefois, les sanctions financières de la Cour des comptes relèvent d’un régime spécifique et ne sont pas considérées comme pénales. Dès lors, les agents concernés ne peuvent pas bénéficier de la protection fonctionnelle de manière automatique. Les agents sont placés dans une situation particulièrement vulnérable en cas de contentieux. Ce manque de garanties pourrait, à terme, nuire à l’attractivité de la fonction publique et freiner l’engagement des cadres dirigeants dans les collectivités territoriales. Dans ce contexte, madame la ministre, pourriez vous nous indiquer quelles mesures sont envisagées afin de mieux encadrer le champ des responsabilités des gestionnaires publics et leur assurer une protection juridique adaptée ? La parole est à Mme la ministre ministre déléguée. Monsieur le sénateur Fabien Genet, je vous remercie d’appeler l’attention du Gouvernement sur l’attente forte des gestionnaires publics sur ce sujet,

Ce texte vise à permettre à l’administration de porter plainte au nom de l’agent victime, à étendre la protection fonctionnelle à titre conservatoire pour les ayants droit de l’agent et à octroyer la protection fonctionnelle à l’agent entendu librement dans le cadre d’une procédure pénale. Par ailleurs, comme vous le rappelez, en l’état actuel du droit, la protection fonctionnelle n’est pas accordée aux agents publics en cas de procédure devant les juridictions financières, dans la mesure où l’agent n’est ni victime d’attaques ni mis en cause dans une procédure civile ou pénale. Le Conseil d’État l’a confirmé dans une décision du 29 janvier 2025, tout en soulignant qu’« il est toujours loisible à l’administration de lui apporter un soutien, notamment par un appui juridique, technique ou humain dans la préparation de sa défense ».

souligne qu’un éventuel élargissement de l’octroi de la protection fonctionnelle en cas de procédure devant les juridictions financières nécessiterait une réflexion approfondie, notamment eu égard aux objectifs mêmes de la réforme visant à renforcer la responsabilité financière des agents publics et aux conséquences en matière budgétaire. Tout en reconnaissant l’attente exprimée de plus en plus fortement sur le terrain face aux mises en cause des gestionnaires publics, le Gouvernement est bien conscient que les contours de cette forme complémentaire de protection requièrent requièrent une expertise pointue. Les services du Premier ministre ont engagé une réflexion sur le sujet et proposeront ultérieurement, en concertation avec la Cour des comptes, une approche adaptée sur ce sujet.

ont poussé les particuliers et les personnes morales à différer leurs projets. J’avais déjà posé cette question en avril 2024, mais je n’avais pas obtenu de réponse du Gouvernement. Or la situation est loin de s’être améliorée Les délais d’instruction des dossiers liés à MaPrimeRénov’ et aux C2E ont été allongés au delà des deux mois promis, augmentant d’autant les délais de paiement. Ces délais allongés sont sans nul doute le résultat de primes complexes, dont les montants et les modes d’attribution sont modifiés tous les deux mois. Documents aléatoires à fournir, manque de formation des instructeurs, rejet du dossier en raison de l’omission du tampon encreur, demande d’attestation d’adressage en complément de la taxe foncière, version obsolète du formulaire manque d’efficience des opérations de contrôle des travaux réalisés sont autant d’exemples kafkaïens qui retardent les délais d’instruction.

dispositif. Dans un contexte de forte demande, marqué par l’élargissement des bénéficiaires en 2021, la réforme des aides en 2024 et la mise en place du régime des services votés en ce début d’année 2025,

au regard des 540 000 dossiers instruits en moyenne chaque année par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Par ailleurs, l’Anah a renforcé de manière significative sa politique de lutte contre la fraude. L’intensification des contrôles a permis de sécuriser le parcours des ménages, mais a pu également provoquer un allongement des délais d’instruction et de traitement des dossiers. Aujourd’hui, l’Anah se mobilise activement pour fluidifier les parcours des usagers, en mettant en place une équipe dédiée aux situations les plus complexes. Les dossiers en difficulté font l’objet d’un suivi individualisé, d’une analyse systématique des difficultés remontées et d’un accompagnement des usagers. L’agence met également en place une d’identification des dossiers en difficulté avant leur signalement et, enfin, une sécurisation globale des plateformes. Je vous confirme donc que le Gouvernement met en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la qualité et la rapidité du traitement et de l’instruction des dossiers.

une couverture nationale par une autorité organisatrice de la mobilité. Elle a offert aux communautés de communes la possibilité d’assumer cette compétence jusqu’au 31 mars 2021. Au delà de cette date, celles qui n’ont pas pris de décision en ce sens ont vu cette compétence automatiquement transférée aux régions. Les choix des communautés de communes ont été contrastés : certaines ont décidé de conserver la compétence « mobilité », tandis que d’autres l’ont laissée à la région. Une nette différence géographique est observée dans les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, le Grand Est et les Hauts de France, plus de 80 % des communautés de communes ont choisi d’exercer cette compétence. En revanche, en Auvergne Rhône Alpes, en Provence Alpes Côte d’Azur et en Nouvelle Aquitaine, elles sont moins de 30 %.

le report des élections municipales, mais aussi la réticence de certaines régions souhaitant garder cette prérogative et un manque de temps pour évaluer les enjeux d’une telle prise de compétence. Une modification de la LOM intercommunale (EPCI) de délibérer de nouveau sur la prise de la compétence « mobilité », en rouvrant au profit des communautés de communes la possibilité d’engager un nouveau travail sur celle ci pendant un temps déterminé suffisamment long pour fixer finement le contenu des services concernés. Il s’agit de permettre aux territoires de se rendre compétents, lorsqu’ils le souhaitent, à leur rythme et selon leurs besoins. Madame la ministre, je souhaiterais connaître la position du Gouvernement sur cette proposition. La parole est à Mme la ministre ministre déléguée. Madame la sénatrice Florence Lassarade, comme vous l’indiquez, en application de l’article 8 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, la délibération de l’organe délibérant des communautés de communes ayant souhaité devenir autorité organisatrice de la mobilité (AOM) devait intervenir avant le 31 mars 2021. À défaut, c’est la région qui devenait AOM sur le ressort territorial de la communauté de communes concernée à compter du 1 juillet 2021. Depuis cette date, une communauté de communes qui n’aurait pas pris la compétence « mobilité » ne peut plus, si sa position évolue, se la voir transférer par la région. Le Gouvernement partage votre constat sur le caractère contrasté des choix effectués par les communautés de communes dans le cadre de la LOM. Les établissements publics de coopération intercommunale qui n’ont pas conservé la compétence « mobilité » se trouvent, en effet, en difficulté lorsque, ultérieurement, ils souhaitent voir se développer une offre de mobilité sur leur territoire. L’outil qu’est la délégation de compétences, même s’il offre une souplesse dans l’exercice des compétences à l’échelon local, ne permet pas toujours de répondre aux enjeux de manière satisfaisante. Rouvrir aux communautés de communes la possibilité de devenir AOM conduirait néanmoins à revenir sur une organisation territoriale de la gouvernance « mobilité » encore trop récente et, par ailleurs, voulue par les acteurs locaux qui ont eu, comme vous le rappeliez, l’opportunité et le temps de choisir. En outre, cela nécessiterait éventuellement de prévoir des transferts de lignes de transport existantes et qui répondent aux besoins des populations en matière de mobilité. Le Gouvernement réfléchit toutefois à la possibilité de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale de délibérer de nouveau sur la prise de la compétence « mobilité », en la rouvrant au profit des communautés de communes. En tout état de cause, cela nécessitera, au préalable, une discussion avec les régions et les EPCI. La parole

beaucoup ont achevé leur développement urbanistique ou disposent d’une configuration spécifique – les espaces constructibles y sont rares, voire inexistants –, elles sont soumises à des obligations chiffrées et à des délais de réalisation inatteignables. Mais ce n’est pas tout ! La crise immobilière qui frappe très durement le secteur vient encore compliquer la situation, laquelle est aggravée par une flambée des coûts de construction, des taux d’intérêt plus élevés, qui freinent les investissements, et une raréfaction marquée des financements publics comme privés. Nombre d’opérateurs se désengagent ainsi purement et simplement de projets immobiliers pourtant largement avancés, certains ayant même déjà obtenu un permis de construire par la collectivité. Dans ce contexte, les objectifs de la période triennale 2023 2026, qui va bientôt s’achever, sont d’ores et déjà compromis et se révèlent, plus encore qu’avant, totalement déconnectés de la réalité au regard de la crise immobilière que je viens d’évoquer.

triennale, dans un contexte de grande tension budgétaire, qui nous concerne tous ? D’une manière plus générale, envisagez vous de faire évoluer cette législation afin de mieux prendre en compte les spécificités territoriales, et ce

près de 50 % de la production de logements sociaux vers les communes aujourd’hui déficitaires, dans un objectif de mixité sociale. Nous restons attachés à l’enjeu essentiel de développement d’une offre sociale équilibrée sur le territoire. La trajectoire de rattrapage a été adaptée en 2022, dans la loi relative D’une part, la révision du mode de calcul des trajectoires a conduit à réduire les objectifs triennaux. D’autre part, la loi 3DS a ouvert la possibilité d’abaisser encore les objectifs dans le cadre des contrats de mixité sociale. Ainsi, sur les 1 153 communes déficitaires à l’échelon national, 353 contrats de mixité sociale ont été signés, dont 187 permettant un abaissement de l’objectif. Les préfets prennent en compte le volontarisme de la commune, tout comme les difficultés qui s’imposent à elle. Ces considérations seront reconduites pour l’analyse du bilan 2023 2025. nous assistons, avec la baisse récente des taux d’intérêt, à une reprise de la construction. Il nous faut amplifier ce rebond pour relancer durablement la construction et la production sociale, notamment dans les communes déficitaires.

chargé des transports. Madame la ministre, j’attire votre attention sur un projet qui suscite une vive inquiétude dans le Val de Marne et dans l’Essonne : le port industriel de Vigneux sur Seine, porté par l’établissement public Haropa Port, placé sous la tutelle de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) du ministère des transports. L’objectif affiché est clair : développer l’axe Seine, renforcer l’activité industrielle et portuaire. Pourtant, sur le terrain, l’opposition est forte. Le maire d’Ablon sur Seine, Éric Grillon, ainsi que de nombreux élus et habitants, dénonce les effets négatifs de ce projet de plateforme multimodale à vocation régionale sur les rives de Vigneux sur Seine et du pont de franchissement entre Vigneux sur Seine et Athis Mons. Trois préoccupations majeures émergent. D’abord, la mobilité. Le réseau routier est déjà saturé. L’implantation de ce port multimodal, couplée à la construction du pont reliant Vigneux à Ablon, risque

à quelques mètres seulement de leurs habitations. Ensuite, l’environnement. Nous parlons ici de l’une des plus belles rives naturelles de la Seine en Île de France. Ce projet entraînera la destruction et l’artificialisation de plus de 50 hectares de zones humides et d’espaces naturels classés, ainsi que la déforestation de 30 hectares en bord de Seine. Enfin, la concertation. Elle est largement insuffisante. Un projet d’une telle ampleur ne saurait être préparé sans un dialogue approfondi avec les élus locaux et les habitants. Madame la ministre, comment le Gouvernement entend il, développement économique et impératifs écologiques ? Peut on envisager de revoir l’ampleur du projet, d’en adapter la conception afin de limiter ses impacts et de préserver cette zone naturelle essentielle à l’environnement ? Surtout, face aux mobilisations citoyennes et à l’inquiétude parfaitement légitime des élus locaux, quelles garanties concrètes le Gouvernement peut il offrir pour assurer une véritable concertation avant d’engager un projet aux conséquences néfastes et irréversibles ? La parole est à Mme la ministre

Haropa Port, le grand port fluviomaritime de l’axe Seine, est en effet propriétaire d’un terrain d’environ 110 hectares sur la commune de Vigneux sur Seine, dans l’Essonne. Si ce terrain avait été acquis dans les années 1990 avec l’objectif d’y développer une plateforme industrielle portuaire sur sa totalité, je peux vous assurer que ce projet initial n’est plus d’actualité. En effet, le nouveau schéma directeur environnemental de la région d’Île de France (Sdrif E), adopté par le conseil régional le 11 septembre 2024, redéfinit complètement l’aménagement de cette zone. Il prévoit désormais une urbanisation à vocation industrielle et multimodale limitée à 35 hectares le long de la voie ferrée, soit moins d’un tiers de la surface initiale. Plus important encore, il garantit la préservation d’une armature verte en bord de Seine sur la majeure partie du terrain. Cette nouvelle orientation pose les bases d’un projet plus équilibré, qui concilie les enjeux de développement économique et de préservation écologique, en phase avec les défis actuels. En ce qui concerne vos interrogations sur la concertation, je peux vous indiquer qu’Haropa Port est actuellement en phase de réflexion préalable. Une fois le nouveau Sdrif E en application, une concertation approfondie sera engagée avec l’ensemble des acteurs du territoire. Cette démarche permettra d’entendre et de prendre en compte les préoccupations légitimes que vous relayez, qu’il s’agisse des impacts sur le cadre de vie, des nuisances potentielles ou des enjeux de circulation.

Rédigée au début des années 1960, la Charte sociale européenne garantit des droits fondamentaux en matière de santé, de logement, d’éducation, d’emploi et de protection sociale. Or, lors de la signature de ce traité international, la France a choisi d’exclure ses territoires ultramarins de son champ d’application. Cette situation perdure depuis plus de soixante Aucune modification n’a été apportée pour inclure nos trois millions de concitoyens ultramarins. Pourtant, l’extension de la portée de ce texte aux territoires ultramarins ne nécessiterait qu’une simple notification adressée par le gouvernement français au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. D’autres pays européens comptant des territoires ultramarins ont fait des choix différents. À titre d’exemple, les Pays Bas appliquent la Charte à la partie néerlandaise de l’île de Saint Martin, alors que la partie française de cette même île en est exclue. La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a qualifié cette situation d’« inacceptable » dans un avis adopté à l’unanimité. En mars 2024, une réclamation collective contre la France a été déposée devant le Comité européen des droits sociaux (CEDS) par plusieurs associations de défense des droits humains. La semaine dernière, le CEDS a jugé irrecevable une réclamation, au motif que la France n’a pas déclaré qu’elle étendait l’application de la Charte aux outre mer. Cette exclusion pose une question fondamentale d’égalité des droits entre les citoyens de l’Hexagone et ceux des outre mer, particulièrement dans un contexte où les spécificités de nos territoires, notamment La Réunion, nécessitent une protection sociale renforcée. Quelles mesures le Gouvernement entend il prendre pour mettre fin à cette discrimination historique et pour étendre enfin l’application de la Charte sociale européenne aux territoires ultramarins ? Il s’agit ainsi de garantir l’égalité des droits pour l’ensemble des citoyens français, quel que soit leur lieu de résidence, à Saint Denis, Cayenne ou Paris.

C’est précisément le sens de l’action du Gouvernement : le budget des outre mer a été revalorisé de 11 % en autorisations d’engagement et de 6 % en crédits de paiement par rapport au budget initial. L’effort total s’élève à près de 25 milliards d’euros, malgré un contexte budgétaire particulièrement contraint. J’ajoute que, si la Charte ne comporte pas d’effet direct, les réclamations ne pouvant être introduites que par des organismes habilités, cette procédure non contraignante contribue, tout comme les voies de recours nationales et internationales déjà existantes, au principe de l’État de droit,

en France et alertait sur une situation inquiétante. Le dernier rapport sur les morts violentes d’enfants au sein des familles date de 2018. Il dénombrait 363 victimes entre 2012 et 2016, soit un décès tous les cinq jours. Ce chiffre alarmant ne reflète qu’une partie du phénomène, car il ne tient compte ni du « chiffre noir » des néonaticides non révélés ni des enfants victimes du syndrome du bébé secoué non diagnostiqué. Des morts sont donc ignorées, faute d’autopsie sur les corps d’enfants présupposés morts naturellement ou accidentellement. Le manque de données fiables, dû à des absences ou à des erreurs de diagnostic, laisse à penser que le nombre de morts d’enfants est en réalité plus important. En 2022, le Gouvernement affichait dans son plan de lutte contre les violences faites aux enfants l’objectif louable de disposer de données en vue d’une meilleure prévention des infanticides. Malheureusement, rien n’a évolué depuis.

ne permettent pas, à ce jour, d’évaluer le nombre d’enfants tués par leurs parents, qu’il s’agisse d’atteintes volontaires à la vie ou de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

directives visant à mieux appréhender et traiter, sur un plan judiciaire, les morts violentes de mineurs liées à une infraction volontaire commise dans la sphère familiale ou institutionnelle. Cette circulaire invite, par ailleurs, les parquets généraux à informer de manière systématique la direction des affaires criminelles et des grâces de la survenance de tels drames, y compris dans les cas de syndrome du bébé secoué ou de mort en lien avec le suicide des parents.

de retenir les éléments pertinents en matière de prévention et de traitement judiciaire de ces drames, afin de les pérenniser et d’identifier les axes d’amélioration à travailler. Cette circulaire encourage aussi la conclusion de partenariats renforcés avec le milieu médical pour favoriser le signalement des morts violentes d’enfants au sein des familles pouvant notamment être en lien avec le syndrome du bébé secoué.

Depuis le 20 février dernier, et pour la première fois sur le territoire français, les personnes dont la garde à vue est prolongée au sein de la compagnie de gendarmerie de Senlis peuvent utiliser une borne de télémédecine si elles souhaitent bénéficier d’une consultation médicale. Ce dispositif avait été rendu possible par la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2027. Ce qui paraissait être une bonne idée à l’époque l’est tout autant aujourd’hui ! En effet, le dispositif permet d’améliorer le quotidien de tous, en particulier celui des forces de l’ordre. forces de l’ordre. Le recours à la téléconsultation médicale pour les personnes placées en garde à vue est une aubaine, et ce d’autant plus pour des territoires ruraux comme l’Oise, qui sont frappés par la désertification médicale et la saturation des services d’urgence hospitaliers. En effet, ce dispositif garantit le droit de toute personne de consulter un médecin dans les meilleurs délais. Il est également – et surtout – utile pour les forces de l’ordre, auxquelles il permet de gagner un temps précieux.

Alors que les bornes de télémédecine apportent une aide précieuse aux gendarmes tout en améliorant les conditions d’accès à la santé des personnes gardées à vue, il est étonnant que ce genre de dispositif n’existe que dans l’Oise, à Senlis. La France, et tout particulièrement les zones rurales, aurait beaucoup à gagner en utilisant de telles bornes. Ma question est simple l’État compte t il étendre le recours à la téléconsultation médicale par les personnes placées en garde à vue ? La parole est à M. le ministre

et par le décret n° 2024 1041 du 18 novembre 2024 relatif aux modalités de réalisation de l’examen médical à distance

par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, et ce même si aucun examen médical n’est intervenu au cours des vingt quatre premières heures. Ces dispositions sont applicables depuis le 21 novembre 2024.

d’une immatriculation délivrée avant 2009, dans un format que les plus anciens d’entre nous ont bien connu. Certaines opérations, telles qu’un changement de titulaire ou d’adresse, nécessitent au préalable de réaliser une conversion qui peut dans certains cas dérouter l’usager. Mais un parcours guidé permet aujourd’hui aux usagers de réaliser ces opérations sur le portail. Près de 10 000 opérations concernant des véhicules de collection ont été réalisées en 2024,

d’un service efficace de soutien aux usagers, notamment au travers de son centre d’appels ; et vous le connaissez bien, madame la sénatrice, puisqu’il est implanté à Charleville Mézières ! Cette agence met tout en œuvre pour réduire les délais d’attente et améliorer la qualité du service qu’elle assure auprès de l’ensemble des usagers.

Jean Verzelen, le Président de la République a annoncé la création de 239 nouvelles brigades de gendarmerie d’ici à 2027. Ainsi, 80 premières brigades ont été créées dans 64 départements métropolitains et 8 départements ou collectivités d’outre mer. Pour 2025, la volonté du Gouvernement est de poursuivre le plan de déploiement de ces nouvelles brigades, bien que le calendrier de création des unités ne soit pas encore totalement arrêté,

Comme vous l’indiquez, trois projets de création de brigades ont été retenus dans votre département : deux brigades fixes, à Saint Gobain et Aubenton, et une brigade mobile, à Neuilly Saint Front. L’État, pleinement conscient des interrogations des élus locaux, veille à accompagner ces projets dans la durée. L’implication des collectivités locales est un facteur clé de réussite pour l’installation de ces brigades.

Vous le savez, ces fermetures suscitent de vives inquiétudes, tant le rôle joué par les femmes et les hommes de ce service public en matière de maintien de l’ordre et de secours aux personnes est important dans nos territoires ruraux comme urbains.

Au regard du contexte international, de la dégradation des finances publiques et de l’annulation de 8 milliards d’euros de crédits, à ce jour, dans le budget pour 2025, pouvez vous m’assurer que ces nouveaux matériels seront bien livrés,

les hélicoptères Écureuil seront progressivement réformés : la manœuvre générale de retrait du service a débuté et devrait être achevée en 2029. Dans ce contexte, la gendarmerie se trouve contrainte de prendre des mesures de gestion. Des sections aériennes seront fermées temporairement, dont celle de Limoges, le temps de conduire les opérations de maintenance obligatoires de garantir au mieux la sécurité des vols et le contrat opérationnel des forces de gendarmerie. Pour remédier à cette situation, des redéploiements de machines entre les sections aériennes permettront dans un premier temps de préserver au mieux leur fonctionnement. Par ailleurs, un renouvellement de la flotte est entrepris pour une parfaite adaptation aux besoins opérationnels. Je vous confirme que seize hélicoptères de nouvelle génération – H160 et H145 D3 – sont commandés pour remplacer les appareils Écureuils réformés. L’affermissement de la tranche conditionnelle du contrat d’acquisition des appareils H145 D3 d’ici à 2027, au profit du ministère de l’intérieur,

En effet, le renouvellement de la flotte est un impératif pour assurer la disponibilité des moyens aériens et leur adéquation aux besoins opérationnels. Sur le terrain, les élus locaux sont très attachés à la gendarmerie,

Aujourd’hui dispersées sur trois sites vétustes et inadaptés, ces infrastructures ne permettent plus aux quatre vingt dix agents de remplir efficacement leurs missions. Problèmes de salubrité, manque d’espace de travail, non conformité aux normes de sécurité incendie et d’accessibilité, stationnement insuffisant : toutes ces contraintes pèsent sur les conditions de travail des policiers et compromettent leur sécurité. Malgré des travaux ponctuels, ces interventions coûteuses ne règlent pas les problèmes structurels. Face à cette situation, le projet de relocalisation dans les anciens locaux de la Banque de France, à Foix, constitue une opportunité unique. Ce bâtiment sécurisé et fonctionnel permettrait de regrouper l’ensemble des services, tout en optimisant les coûts à long terme. Ce bâtiment, de nouveau disponible à la vente, représente une opportunité qu’il convient de saisir sans tarder. Un retard dans la prise de décision risquerait de compromettre le projet, au détriment des agents et des habitants du département de l’Ariège. Alors que ce projet bénéficie d’un large soutien local, je souhaite savoir si l’État compte acheter dès cette année ces locaux et engager rapidement des travaux, afin de permettre aux agents de la police nationale de l’Ariège d’accomplir leurs missions dans des conditions optimales.

Au début de l’année 2024, le ministre de l’intérieur a passé une commande globale de quarante deux hélicoptères, dont six au bénéfice des forces aériennes de la gendarmerie nationale, auxquelles un premier appareil a été livré en novembre dernier. La section aérienne de gendarmerie de Briançon possède depuis 2008 un appareil Écureuil 145, dont l’usage, du fait de ses caractéristiques techniques limitées, est de moins en moins opérant. Le peloton est aujourd’hui la deuxième de France. Il réalise plus de mille missions aériennes chaque année, dont certaines demandent un grand professionnalisme et du matériel performant. Je pense ainsi à l’opération du 24 décembre dernier, l’évacuation de 240 skieurs bloqués sur un télésiège en panne à la station de Superdévoluy dans le département des Hautes Alpes. Vous l’aurez compris, la livraison de ce nouvel hélicoptère H145, plus puissant que la machine actuelle, est nécessaire pour élargir le spectre des opérations de secours réalisables. En effet, son moteur, beaucoup plus puissant que celui de l’Écureuil, autorise, par exemple, l’emport d’un nombre supérieur de personnels, mais aussi de davantage de matériel.

la flotte aérienne de la gendarmerie nationale est vieillissante : elle requiert une vigilance particulière en termes de maintenance et nécessite un renouvellement significatif. Un marché d’acquisition de H145 D3 a été notifié. Il comprend une tranche ferme de six appareils et une tranche complémentaire de vingt deux appareils. Sur les six premiers hélicoptères,

Les quatre autres seront répartis de la manière suivante : le premier sera affecté à la section aérienne de gendarmerie de Chamonix en 2026 un autre, livré en 2027, sera positionné au centre national d’instruction ; les deux derniers seront affectés à la section aérienne de Cayenne à la fin 2027 et au début 2028. Il n’est donc pas prévu, pour le moment, de doter la section aérienne de gendarmerie de Briançon d’un H145 D3 avant 2028, si ce n’est ponctuellement. Convaincus de la nécessité de renouveler le parc des EC145, en particulier dans les unités de haute montagne telles que Briançon, Briançon, où les conditions de vol et d’engagement opérationnel peuvent être particulièrement difficiles, nous travaillons à ce que la tranche complémentaire des vingt deux H145 D3 soit affermie avant 2027. Le ministre de l’intérieur me charge de vous indiquer que la demande de la section aérienne de gendarmerie de Briançon sera alors étudiée en priorité, en raison de l’activité opérationnelle intense que vous avez, à juste titre, évoquée. chers collègues,

de nuit qui ne sont en rien des petits commerces de proximité. Ces établissements, particulièrement concentrés dans le nord est de la ville, sont bien souvent les vitrines d’un système de blanchiment d’argent, au service du crime organisé. Ils alimentent l’insécurité, entraînent des nuisances permanentes et fragilisent notre tissu économique local en instaurant une concurrence déloyale avec le commerce traditionnel. Pourtant, que fait la maire de Paris ? Rien ! Pis, elle ferme les yeux. Par dogmatisme ou par lâcheté, Mme Hidalgo refuse d’agir. Elle laisse les réseaux criminels s’installer, prospérer, s’enraciner dans nos quartiers. La proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic prévoit notamment la possibilité, pour un maire, de demander la fermeture administrative d’un commerce suspecté de blanchiment.

Sur instruction du ministre, le préfet de police de Paris a déjà mis au jour du travail dissimulé, des emplois d’étrangers sans titre et de la fraude fiscale. Il continuera son action pour déposséder les délinquants de leur patrimoine, saisir leurs biens et ceux de leur entourage. Le texte sur le narcotrafic l’y aidera. Madame la sénatrice, vous pouvez compter sur l’engagement du ministre de l’intérieur et de l’ensemble des forces de l’ordre pour lutter contre le blanchiment et le narcotrafic en général. Nous en

Merci